A1.2, nous proposons que notre fiscalité cesse d’être mise au service de la subvention des véhicules les plus lourds et les plus polluants.

au titre de l’emploi d’un salarié à domicile. Avec 6,17 milliards d’euros estimés pour 2024, le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est la deuxième dépense fiscale la plus coûteuse pour les finances publiques. Elle est la première concernant l’impôt sur le revenu. Son coût n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années, passant de 4,85 milliards d’euros à 6,17 milliards d’euros en cinq ans. La loi de finances pour 2023 oblige le contribuable à renseigner, dans sa déclaration annuelle de revenus, les activités au titre desquelles il sollicite le bénéfice de ce crédit Cette évolution législative permet de constater que 50,4 % de la dépense fiscale a été consacrée à l’entretien de la maison et aux travaux ménagers en 2022, soit près de 3 milliards d’euros d’après la prévision du crédit d’impôt en 2023. du crédit d’impôt prévu pour des frais engagés pour la garde, l’accompagnement d’enfants, l’assistance et l’aide aux personnes âgées ou handicapées se comprend aisément, il est toutefois moins défendable quand il s’agit de financer l’entretien de la maison et les travaux ménagers pour des personnes valides. Néanmoins, il constitue aussi un instrument de lutte contre le travail non déclaré. Aussi, dans un souci de concilier la lutte contre le travail dissimulé et le redressement des comptes publics, amendement tend à instaurer un taux dégressif pour cette activité. Il demeurerait inchangé à hauteur de 50 % jusqu’au sixième décile de revenu inclus, avant de passer à 30 % pour les septième et huitième déciles, puis à 10 % pour les deux derniers déciles. Quel

et dans lequel elle verra comme un prolongement de son propre domicile. Ainsi, cet amendement vise à étendre aux structures d’accueil non médicalisé le crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile

plus grand nombre de personnes âgées, en particulier celles ne disposant que d’un revenu moyen ou faible. Dès lors, la meilleure solution de financement est la défiscalisation des frais d’accueil des bénéficiaires.

auquel la personne âgée peut aisément faire appel et dans lequel elle verra comme un prolongement de son propre domicile. Ainsi, cet amendement vise à étendre aux structures d’accueil non médicalisé le crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile à une association agréée ou à un organisme habilité

par des particuliers employeurs, et de l’autre, celles qui sont versées à des organismes de services à la personne. Cet amendement présente

qui explique que le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire soit particulièrement important cette année. Les finances des organismes caritatifs sont sous pression. L’ensemble de ces organismes, comme les banques alimentaires, mais aussi les Restos du Cœur,

d’impôt concerne seulement les bénévoles imposables. Or les bénévoles non imposables, au même titre que ceux qui sont imposables, donnent de leur temps et engagent des dépenses afin d’œuvrer à améliorer le quotidien des personnes.

Les bénévoles non imposables, qui disposent de plus faibles revenus, font face, comme l’ensemble de la population, à une inflation croissante. Cet amendement vise à remédier à l’inégalité de traitement vécue par les bénévoles non imposables. Cet amendement est soutenu par le Mouvement associatif, dont le Secours catholique, qui rappelait l’urgence d’une telle mesure lors de sa quatrième rencontre du groupe parlementaire du 15 novembre, du fait du coût dissuasif des frais de déplacement de ses bénévoles en milieu rural.

le Sénat examinera une proposition de loi présentée par notre groupe, visant à instaurer une allocation d’autonomie universelle d’étude pour tous les jeunes de 18 à 25 ans. Il y a quelques jours, un représentant des Restos du Cœur expliquait que les jeunes de moins de 25 ans représentent désormais la moitié des bénéficiaires Face à cette situation critique, une réforme structurelle de la politique de soutien à la jeunesse nous apparaît absolument prioritaire, alors que les dispositifs qui lui sont adressés se fondent trop souvent sur la politique de soutien à la famille. Il paraît invraisemblable que les aides fiscales destinées aux jeunes de 18 ans transitent encore par le foyer fiscal familial. Je pense à la demi part de quotient familial ou encore à la réduction d’impôt pour un jeune majeur scolarisé dans le supérieur.

font l’objet d’un cofinancement par l’État, les collectivités territoriales, ainsi que par l’industriel à l’origine du risque, laissant un reste à charge de 10 pour les particuliers. Depuis 2013, ces travaux prescrits font l’objet d’un double plafond : leur montant ne peut excéder 20 000 euros ou 10 % de la valeur vénale du bien. Ce plafond n’a pas été révisé depuis 2013. Pourtant, durant la même période, les prix du bâtiment ont augmenté d’environ 25 %. Cet amendement vise donc à augmenter le montant maximal des travaux prescrits, en le faisant passer de 20 000 euros Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que le relèvement de ce plafond entraîne uniquement une augmentation du crédit d’impôt de l’État. Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs je vous remercie

en faisant du taux d’imposition individualisé le taux applicable de droit commun. Cette mesure a d’ailleurs été annoncée par la Première ministre le 8 mars

ou accessoires. Ces écarts s’invitent dans le rapport au travail, si bien que le recours au temps partiel est près de quatre fois supérieur pour les femmes, de

diminuer de 13 points. En conséquence, « le revenu des femmes est davantage taxé qu’il ne le serait en l’absence d’imposition commune, ce qui a un effet dissuasif sur le travail féminin et crée de véritables trappes à inactivité ».

La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote. opportun, qui constitue une avancée en matière d’individualisation de l’impôt sur le revenu. Le groupe socialiste lui apportera donc tout son soutien. La parole

Le droit à l’information est d’ailleurs protégé constitutionnellement depuis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le premier rempart, c’est la diffusion de vraies informations la publication de faits vérifiés par des journalistes respectant les règles déontologiques dans les journaux ou les sites de référence identifiés comme tels par les citoyens. Depuis plusieurs années, le secteur de la presse connaît une crise structurelle liée à la chute des abonnements et au report des annonceurs vers internet au profit des Gafam

Pour autant, nous considérons que ce n’est pas suffisant. Le réflexe citoyen de l’abonnement à des titres de presse est en recul, ce qui rend les journaux plus dépendants des autres sources de financement que sont la publicité et les aides à la presse. Alors que plus de 53 % des citoyens expriment une défiance envers les journalistes, au motif qu’ils seraient trop dépendants des pouvoirs économiques et politiques, il importe de raviver le réflexe de l’abonnement chez tous nos concitoyens.

années de mariage. Le droit prévoit que la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée en cas de disproportion entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

dès lors que, pendant leur période d’imposition commune, les conjoints partagent le même train de vie et déclarent ensemble leurs revenus. Le manquement aux obligations déclaratives concerne, au moins indirectement, les deux conjoints, qui établissent la déclaration commune.

par la prise en compte des difficultés financières du demandeur. En créant un nouveau motif de décharge, qui n’est pas fondé sur la situation matérielle du demandeur, le dispositif proposé risque de générer une rupture d’égalité injustifiée devant la charge fiscale. Enfin, ce nouveau motif crée un risque de contournement et ouvre une voie de soustraction à l’impôt, ce qui pourrait porter atteinte à la garantie de recouvrement des créances fiscales,

Cet amendement vise donc à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur en excluant sa résidence principale, lorsqu’il en est propriétaire ou qu’il détient sur elle un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs ainsi que le patrimoine qu’il a reçu par donation ou succession.

Ces amendements ont pour objet de préciser notamment les critères d’examen des demandes de décharge de responsabilité solidaire formulées par les anciens conjoints. Il s’agit également d’encadrer les critères d’appréciation de la situation patrimoniale

vise à soumettre à un même taux d’imposition les transferts fonciers entre personnes physiques et les cessions de parts sociales, actuellement favorisées fiscalement. À cette fin, nous proposons de porter les droits d’enregistrement à 5 % pour les cessions de participations

objet d’asseoir les droits d’enregistrement sur la valeur réelle des seuls immeubles et droits immobiliers détenus par lesdites personnes morales, sans en déduire les dettes contractées. Il s’agit de rétablir une égalité avec toutes celles et ceux qui s’acquittent simplement des droits de mutation

la cession des titres de la société a pour objet de conférer à la société bénéficiaire la majorité des droits sur un actif immobilier, afin d’éviter que les communes ne soient privées de leur droit de préemption.

Il faut entrer dans les détails techniques – où je suis sûr que vous allez me supplanter. Vous le savez, le régime d’imposition des cessions de parts sociales d’une SCI, par exemple, conduit à imposer ce type de cession de façon bien moins importante que dans le cadre d’une vente entre particuliers.

avec des barèmes hétérogènes en fonction de la date d’ouverture du contrat et des âges auxquels ont été effectués les versements. De fait, la transmission de patrimoine l’assurance vie a connu ces dernières décennies une très forte augmentation. Selon la Fédération française de l’assurance,

Pour plus de justice fiscale, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires estime important d’abroger l’exonération spécifique à la transmission d’un contrat d’assurance vie en la faisant entrer dans le barème global des DMTG.

que cette mesure vient limiter le risque d’optimisation fiscale.

du conjoint et de certains de leurs enfants. Cet abattement, d’application automatique pour déterminer les droits de succession, peut s’avérer pénalisant en termes de plus values. Ainsi, en cas de revente du bien rapidement après le décès, l’application de l’abattement de 20 conduit les héritiers, qui ne peuvent profiter de l’exonération pour résidence principale, à payer un impôt sur la plus value immobilière plus important que l’économie réalisée sur les droits de succession. À défaut d’autres cas d’exonération, l’impôt sur la plus value est dû, alors même que le logement serait vendu à un prix égal à la valeur vénale réelle au jour de la succession. Pour des raisons de justice et de souplesse fiscales, le présent amendement a pour objet de rendre optionnelle l’application de l’abattement de 20 %.

l’avis du Gouvernement ? Monsieur le sénateur, la condition que l’activité de holding animatrice de groupe constitue l’activité principale de la société résulte de la jurisprudence

en remplaçant le taux d’exonération par un abattement fixe de 2 millions d’euros. Cela reviendrait purement et simplement à plafonner l’avantage fiscal

Quel est l’avis de la commission ?

tant en cas d’imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU) qu’en cas d’imposition au barème progressif. Toutefois, seules les plus values sur les titres détenus par le dirigeant bénéficient de l’abattement. Les plus values

question des stocks, l’administration fiscale a précisé, dans ses commentaires, qu’ils n’étaient pris en compte que lorsqu’ils contribuaient à la valorisation des éléments transmis, ce qui s’inscrit dans la logique même du dispositif.

Dès lors, afin d’encourager le renouvellement des générations, cet amendement vise à accorder au cédant le bénéfice du dispositif d’exonération lorsque ce dernier accepte de fractionner son exploitation en vue d’une cession répartie entre différents repreneurs, tous jeunes agriculteurs.

au détriment des paysannes et paysans et du dynamisme de nos campagnes. Nous proposons de porter les droits d’enregistrement à 5 % pour les cessions de participation dans des personnes morales exerçant une activité agricole, à titre principal ou accessoire. Pour ne pas pénaliser les exploitations familiales, un droit d’enregistrement fixe de 125 euros serait maintenu pour les associés exploitants des groupements sous réserve qu’ils contrôlent après la cession une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne, fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Un droit fixe de 125 euros serait également maintenu pour les cessions de gré à gré des parts de groupements fonciers agricoles

(FNSafer), les lots acquis par les sociétés sont en général « 27 % plus grands et 5,2 fois plus onéreux que ceux acquis par des personnes physiques ». Cette dynamique alimente la flambée des prix qui peut être observée dans certaines localités également la raréfaction des terres disponibles à l’installation. La France a perdu 100 000 exploitations en dix ans. À l’horizon 2030, 50 % des paysans partiront à la retraite.

d’autant que, durant la dernière campagne présidentielle, le Président de la République s’était lui même prononcé pour une baisse de la fiscalité sur les successions et les donations. Les amendements

Alors que les héritiers sont souvent les premiers bénéficiaires du capital social et culturel de leurs parents, l’exonération actuelle de 100 000 euros tous les quinze ans permet de se soustraire une fois de plus à la contribution à la solidarité nationale. Nous proposons de faire disparaître cette règle

du Sénat sur cet amendement. La loi du 22 juillet 2023 a permis de mettre en place une procédure administrative destinée à accélérer la restitution de biens spoliés dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945. Notre ancienne collègue Corinne Bouchoux avait souligné toutes les entraves aux restitutions liées aux limites des dispositifs établis par l’ordonnance du 21 avril 1945 modifiée par la suite. À raison, le présent article, issu d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale, prévoit une exonération des droits de mutation par décès pour ces biens spoliés qui renvoient à des histoires familiales particulièrement douloureuses.

Cet amendement vise surtout à s’assurer que la rédaction couvre l’ensemble des situations de restitution, dès lors que l’article ne vise pas l’ordonnance du 21 avril 1945.